La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 26 février 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. Mes chers collègues, par lettre en date du 28 février, le Gouvernement, sur proposition du président du Sénat, demande l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 4 mars, le soir, d'un débat sur les mesures de santé publique prises face aux risques d'une épidémie de coronavirus Covid-19 en France. En conséquence, la suite du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, initialement prévue le même jour l'après-midi et le soir, est reportée au jeudi 5 mars, matin et après-midi. Acte est donné de cette demande. Dans l'organisation du débat, à la suite de l'intervention liminaire du Gouvernement, la commission des affaires sociales disposerait d'un temps de huit minutes ; puis, la parole serait donnée à un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun, ainsi qu'à un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes ; enfin, se tiendrait une séquence de quinze questions-réponses. Le délai limite d'inscription des orateurs des groupes serait fixé à, aujourd'hui, dix-sept heures.

de rappeler que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Inde, qui est, quant à elle, le neuvième partenaire commercial de l'Union. Le volume total des échanges de biens et services est en constante augmentation. Il en va de même pour le volume global des flux et des stocks d'investissements directs étrangers. Par ailleurs, environ 6 000 entreprises de l'Union européenne sont implantées en Inde et fournissent 1,2 million d'emplois.

la Commission européenne a lancé en 2007- voilà treize ans -des négociations en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange. Ces négociations ont

Il ne faudrait pas que l'Union européenne soit en quelque sorte doublée par les États-Unis, mais, contrairement à ceux-ci, elle n'a toujours pas renoué le dialogue avec l'Inde. Lors du dernier sommet

sont toutes deux très actives pour conforter ce lien, qui se traduit aussi en termes d'investissements. En effet, la France est le dixième investisseur étranger en Inde, avec un stock d'investissements de 9 milliards d'euros ; près de 550

que nous puissions adopter un programme de travail pour les cinq prochaines années. Ces sujets commerciaux, comme je l'ai dit au ministre du commerce, doivent également figurer en haut de l'agenda compte tenu des intérêts mutuels.

Ces praticiens exercent dans nos hôpitaux comme palliatif au manque de professionnels dans les établissements de santé des zones sous-denses, parfois de manière illégale, le plus souvent dans une grande précarité, la loi ne reconnaissant ni leur formation ni leurs compétences.

le débat sur le statut de ces praticiens- souvent français -, pas plus qu'elle n'a réglé le devenir de leurs carrières, en reliant par exemple ces questions à l'exercice de leurs compétences en dehors de l'hôpital, dans un autre cadre en tension de notre médecine française : les déserts médicaux. Or, pour certains élus locaux, installer des médecins généralistes dans leur bassin de vie est une priorité. Ces praticiens diplômés pourraient alors mener des carrières mieux rémunérées, moins précaires et plus utiles dans ces territoires où la densité médicale est faible et la mortalité plus élevée que la moyenne nationale. Des mesures d'incitation à l'installation dans de tels bassins de vie pourraient constituer une solution à moyen terme, dans l'attente des répercussions de la suppression du sur la population médicale. alors que la question de la situation de ces praticiens devient une arlésienne pour laquelle sont régulièrement prises des dispositions provisoires, quand et comment une réponse claire pourra-t-elle leur être apportée, alors même que, sous réserve des contrôles de qualification nécessaires,

précise. Vous l'avez rappelé, la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a mis en place de nouvelles mesures visant à permettre aux praticiens à diplôme hors Union européenne, les fameux Padhue, qui exercent en France sans avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances ou à tout autre dispositif d'autorisation d'exercice, de construire un véritable projet professionnel tout en garantissant la sécurité des soins que nous devons à nos concitoyens. Souvent placés dans des situations professionnelles précaires- vous l'avez indiqué -, les professionnels déjà en exercice pourront, sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité fixées par la loi, faire valoir et faire reconnaître leur expérience professionnelle et leurs compétences et se voir prescrire, si besoin, un « parcours de consolidation des compétences », qui sera réalisé au sein de l'une des structures agréées pour la formation des étudiants de troisième cycle, et ce en vue d'obtenir le plein exercice en France. La loi de 2019 a également rénové et assoupli le dispositif d'autorisation d'exercice de droit commun du concours annuel de la liste A à compter de l'année 2020. remplace le recrutement direct de gré à gré par les établissements des praticiens lauréats des épreuves annuelles de vérification des connaissances par un dispositif d'affectation ministérielle sur la base d'un recensement effectué par les agences régionales de santé, tenant justement compte des besoins des territoires et des demandes exprimées par les établissements de santé. Par ailleurs, c'est également au travers du dispositif rénové du contrat d'engagement de service public (CESP), allocation versée aux étudiants en médecine en contrepartie d'une installation dans une zone sous-dense,

Il reste en effet aujourd'hui très complexe, pour nombre de ces victimes, d'obtenir la reconnaissance et la réparation de leur préjudice. Celles-ci doivent remplir de nombreuses conditions, à leurs frais, pour engager une procédure contentieuse devant les tribunaux qui ait quelque chance de succès : il faut agir avant que l'action ne soit plus recevable, démontrer qu'un lien de causalité entre une prise de médicament et la survenue de l'effet indésirable est à l'origine du dommage et parvenir à établir les responsabilités.

pour la plupart d'entre elles, c'est impossible : on peut considérer que seulement 1 % des personnes concernées ont pu agir devant la justice. se tourner vers l'Oniam, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Cependant, cette voie dite « amiable » est souvent une impasse pour les victimes de médicaments autres que le Benfluorex et le Valproate de sodium, notamment du fait du degré de gravité requis pour solliciter une indemnisation. Beaucoup de victimes sont démunies.

2016 est un premier élément de réponse, dont il conviendra, je vous le concède, d'évaluer la pertinence sur le long terme. Les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité pour les victimes de demander leur indemnisation par l'exploitant du produit dans le cadre du dispositif de règlement amiable

Le cas échéant, l'Oniam assure une indemnisation sur fonds publics, au titre de la solidarité nationale, si l'exploitant du produit refuse d'assumer ses responsabilités. Si ce dispositif constitue un niveau de réponse adapté face aux accidents médicamenteux individuels ou de faible ampleur, les pouvoirs publics n'ont pas manqué de l'adapter dans les hypothèses d'accidents sériels de plus grande ampleur, tels que ceux que vous avez évoqués. Ainsi, pour les accidents liés aux médicaments commercialisés sous les noms de Mediator ou de Dépakine, l'État a pris l'initiative de mettre en place, en 2011, puis en 2016, des dispositifs spécifiques d'indemnisation au sein de l'Oniam. On peut également noter que, s'agissant du médicament commercialisé sous le nom d'Androcur, les commissions de conciliation et d'indemnisation saisies dans le cadre du dispositif de droit commun de l'Oniam ont adopté une méthodologie commune, qui permettra d'apporter une réponse homogène et équitable sur l'ensemble du territoire. Dans ces conditions, la mise en Dans ces conditions, la mise en place d'un fonds d'indemnisation des accidents médicamenteux, qui, en tout état de cause, ne pourrait indemniser les effets indésirables des produits en dehors de toute recherche de responsabilité en matière de produits défectueux, ne nous apparaît pas

constitue un outil adapté et pertinent, qui peut être ajusté au besoin, comme cela a été le cas par le passé. La parole

Ce ratio est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Cela a conduit l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire à réaliser plusieurs études, ainsi que des investigations environnementales. En novembre dernier, l'Agence nationale de santé publique a présenté les résultats de l'étude épidémiologique menée depuis mars 2019. Ces résultats confirment le nombre de cancers supérieurs à la moyenne nationale sur les sept communes concernées, mais indiquent qu'aucune cause susceptible d'expliciter ces résultats Le 18 novembre, Santé publique France a conclu à la présence d'un regroupement spatio-temporel sans cause commune identifiée. L'Agence a alors annoncé sa décision de ne pas poursuivre d'investigations et de prélèvements environnementaux supplémentaires. Cette décision est inadmissible. Elle est vécue comme un véritable abandon de la puissance publique. Les familles reprochent notamment à l'ARS l'obsolescence de la méthodologie, focalisée sur la recherche de valeurs de toxicité aiguë, alors qu'elles estiment qu'il faudrait étudier une toxicité chronique et des effets « cocktail ». Des études environnementales complémentaires seraient également nécessaires. Les parents des enfants malades, devant le manque de soutien du Gouvernement, envisagent même de se cotiser pour financer ces études. Cela n'est pas admissible dans une République où la solidarité nationale s'impose à tous.

... Cependant, vous le savez, ces investigations n'ont pas permis d'identifier de cause commune. En complément de l'enquête épidémiologique, des investigations environnementales ont été conduites par l'ARS et la Dreal des Pays de la Loire- avec l'appui des agences nationales -pour repérer d'éventuels dépassements des valeurs de référence. Des centaines de prélèvements et de mesures ont été réalisées concernant l'eau, l'air, les sols, les champs électromagnétiques, les rayonnements ionisants ... Ces investigations se poursuivront jusqu'à leur terme. terme. Si cela se révélait nécessaire, des mesures seront prises pour protéger les personnes concernées. Ce type de pose de nombreuses questions, dont beaucoup restent à ce jour, en l'état actuel des connaissances, sans réponse. Il faut donc poursuivre et amplifier la recherche sur les causes des cancers pédiatriques, afin de permettre, demain, une meilleure compréhension et donc une amélioration de leur prévention dans votre territoire et bien au-delà. Santé publique France contribue à l'avancée des connaissances, à travers des études épidémiologiques de grande ampleur. C'est également le but de la dédiée à la recherche fondamentale en cancérologie pédiatrique que pilote l'INCa. Enfin, les débats qui ont entouré ces investigations ont souligné, à juste titre, la nécessité d'agir par la prévention et le plus précocement possible pour améliorer les milieux de vie. L'agence régionale de santé des Pays de la Loire a ainsi proposé d'engager des actions de prévention pour améliorer la qualité de vie des habitants de Sainte-Pazanne et des communes environnantes : dépistage du risque radon, réduction des expositions aux pesticides, urbanisme favorable à la santé, lutte contre l'habitat insalubre, amélioration de la qualité de l'air intérieur Cette mobilisation pourra notamment se concrétiser par la signature prochaine d'un contrat local de santé entre les élus locaux concernés, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire et les autres services de l'État. Je ne doute pas, monsieur le sénateur, que vous serez associé à ces travaux.

Alors que la convention nationale 2016-2021 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie a fixé la nomenclature des dispositifs mis en oeuvre pour inciter les professionnels de santé à s'installer en zone sous-dense, il apparaît qu'un certain nombre d'élus locaux constatent un phénomène qualifié de « nomadisme médical se caractérise par le fait, pour un professionnel de santé, de s'installer sur un autre territoire au terme de la courte période ouvrant droit aux financements prévus par ces dispositifs conventionnés, pour pouvoir bénéficier de nouveaux financements, et ce alors même que ces mesures financières incitatives sont souvent accompagnées d'investissements particulièrement lourds pour certaines communes. Nonobstant le fait que l'esprit même de ces aides serait ainsi détourné, ce phénomène est de nature à fragiliser un peu plus la crédibilité du principe de libre installation qui caractérise l'exercice de la médecine libérale, déjà régulièrement interrogé par les pouvoirs publics au travers de diverses propositions visant à le supprimer ou, pour le moins, à le nuancer. Aussi, je souhaiterais savoir s'il existe un outil spécifique de contrôle entre les ARS afin d'éviter ce phénomène et de connaître les limites fixées à la possibilité d'une cumulation dans le temps de ces différents dispositifs. La parole

contrat d'aide à l'installation des médecins, un contrat de transition pour les médecins, un contrat de solidarité territoriale médecin et, enfin, un contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins. Ces dispositifs, gérés par l'assurance maladie, proposent des aides à l'installation aux médecins souhaitant exercer dans les zones sous-denses, ainsi que des mesures visant à faciliter leur bonne coordination et leur stabilisation sur ces territoires. Par ailleurs, des contrats gérés par les agences régionales de santé ont vocation à garantir une rémunération minimale

en un contrat unique appelé « contrat de début d'exercice », ouvert à l'ensemble des médecins s'installant dans une zone sous-dense, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, ainsi qu'aux remplaçants exerçant dans ces territoires.

En cas de résiliation anticipée, sachez que les sommes perçues devront être restituées au prorata de la durée restant à couvrir. Un outil a par ailleurs été développé par l'assurance maladie, permettant aux caisses de détecter d'éventuels cumuls de contrats pour un même médecin. Afin d'informer les élus territoriaux sur les aides versées par l'assurance maladie et par l'État, les services du ministère ont rédigé un guide pratique, intitulé et publié en novembre 2019. Il permet aux collectivités territoriales de cibler au mieux leurs dispositifs d'aide à destination des médecins et d'éviter ainsi

santé. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite vous interpeller au sujet de la rédaction de l'avis d'arrêt de travail pour congé maladie dans le cas où le patient est un élu local. De nombreux élus se voient réclamer le remboursement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie, en raison de l'exercice de leur mandat pendant leur arrêt. Très peu d'entre eux savent qu'ils doivent solliciter une autorisation d'exercer une fonction élective durant le congé maladie. Or de nombreuses maladies, surtout en cas de longue maladie, peuvent contraindre à un arrêt de travail sans empêcher un élu de passer une heure par jour à la mairie. a publié un document informant les élus de cette disposition. Cependant, tous n'ont pas eu accès à l'information. Pis, et c'est le cas dans mon département, ceux qui se mettent en conformité lors du renouvellement de l'arrêt maladie après avoir lu cette publication se voient redressés pour les arrêts antérieurs. Ces élus de bonne foi ne peuvent se prévaloir du droit à l'erreur introduite dans la loi pour un État au service d'une société de confiance, car c'est le médecin

signaler que le praticien doit expressément autoriser les activités d'élu. Une case pourrait également apparaître sur le document Cerfa, spécifiant les activités autorisées pendant l'arrêt de travail. Cette solution serait le meilleur moyen pour informer praticiens et élus locaux de l'obligation.

bien compréhensible, de préservation de la santé du patient et de son entourage. Si l'élu local continue d'exercer son mandat, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer les indemnités journalières

Le médecin est le seul apte à estimer, sur la base de l'examen individuel, si cette activité est compatible avec l'état de santé du patient, disposant de la faculté d'autoriser toute activité qu'il juge possible. Nous serons tous d'accord pour le dire : il faut qu'il en reste ainsi C'est d'ailleurs le sens des nouvelles dispositions introduites par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique en son article 103, qui précise que les élus locaux peuvent continuer à exercer leur activité en tant qu'élu, sous réserve de l'accord formel de leur médecin.

des informations pratiques aux élus locaux sur cette faculté en cas d'arrêt de travail. Cette page mentionne notamment la nécessité d'être autorisé par le médecin à exercer son mandat pour percevoir des indemnités

de travail. Le formulaire d'avis d'arrêt de travail, qui est en cours d'évolution, pourrait en effet faire apparaître distinctement la possibilité d'exercer une activité sur autorisation expresse du médecin dans une case spécifique,

Grâce aux efforts conjugués des équipes du pôle Femme Mère Enfant du CHM, des pédiatres de la clinique du Tertre Rouge, des pédiatres quittant le CHM ou encore des CHU d'Angers et de Nantes, le planning médical est aujourd'hui sécurisé jusqu'en novembre prochain. La maternité du Mans a donc, pour le moment, préservé son niveau 3, qui lui permet d'accueillir les nouveau-nés et leur mère venus des départements voisins. Je tiens ici à saluer la solidarité des médecins et la coopération régionale qu'a su faciliter le directeur général du CHM, M. Olivier Bossard, ainsi que ses équipes. Cette solidarité interdépartementale est sans doute une des réponses à apporter pour endiguer la désertification médicale, même si elle ne peut être suffisante en soi. En effet, l'équilibre demeure fragile, et le risque de déclassement du CHM n'est pas encore totalement écarté.

Le 14 février dernier, les chefs de service vous ont appelé à une révision profonde du mode de financement, afin d'inciter à la pertinence des soins, plutôt qu'au développement des seules activités rentables pour l'établissement. Même si une dynamique positive est lancée pour le maintien d'un service de néonatologie performant au Mans, je souhaite connaître l'accompagnement dont bénéficiera le CHM

Les responsables du centre ont pris toute une série de mesures touchant à l'organisation interne et aux activités du service : recherche active de praticiens avec le soutien de l'agence régionale de santé ; fermeture des quatre lits de réanimation pédiatrique pour sauvegarder la réanimation néonatale,

conditions de sécurité et les protocoles de prises en charge sont assurés en liaison très étroite avec le CHU d'Angers et tous les autres établissements concernés. Une coopération a été établie entre le centre hospitalier du Mans et la clinique du Tertre Rouge, disposant d'une autorisation de soins intensifs. Les réanimateurs pédiatres de cet établissement viendront assurer des gardes au centre hospitalier afin de compléter l'équipe. Une réorganisation a été mise en oeuvre pour permettre à l'équipe restante de se concentrer sur les prises en charge intensives. L'ARS a réuni les différents acteurs- CHU de Tours, Angers, Nantes et la clinique du Tertre Rouge au Mans -à plusieurs reprises. Les CHU de Tours et d'Angers se sont ainsi engagés à mettre en place, dès le mois de novembre, des postes d'assistants partagés avec le centre hospitalier du Mans. Les appuis trouvés au sein de l'équipe de pédiatrie du Mans, avec les pédiatres de la clinique du Tertre Rouge, avec les CHU d'Angers et de Nantes permettent de consolider le tableau de gardes jusqu'en novembre 2020 et de maintenir les activités, hormis la réanimation pédiatrique. Le centre hospitalier du Mans poursuit sa recherche de médecins pédiatres

Encore moins si l'article 36 du projet de loi ASAP, en cours de discussion, est voté, puisqu'il prévoit d'allonger encore d'un an le délai d'habilitation établi par la loi de 2018. C'est une vraie course de lenteur ! En attendant, En attendant, les problèmes que ces ordonnances sont censées régler demeurent, notamment ceux que pose aux élus des petites communes l'inadaptation de la législation et de la réglementation relatives aux crèches et à leur manque de moyens. Ces élus sont dans l'impossibilité de répondre aux attentes des parents, particulièrement de ceux qui travaillent. Sont très attendues les possibilités, évoquées lors des consultations ayant précédé la demande d'habilitation, à l'obligation générale d'un espace minimum de 7,5 mètres carrés par enfant et d'assouplissement des modalités d'accueil en surnombre, la même qualité d'accueil étant par ailleurs garantie. Monsieur le secrétaire d'État, peut-on espérer que les élus et les parents des petites collectivités ne seront pas déçus ? Si oui, peuvent-ils, en attendant le texte définitif- j'insiste particulièrement sur ce point -, bénéficier de dérogations qui leur permettraient

pouvant concourir au développement et au maintien de l'offre d'accueil du jeune enfant. Une concertation s'est tenue, de septembre 2018 à septembre 2019, avec l'ensemble des parties prenantes. Elle a fait l'objet d'un rapport rendu public en décembre 2019, rapport que vous avez

Parmi les mesures envisagées, se trouvent la simplification du pilotage local de la politique d'accueil du jeune enfant et la transformation des relais d'assistants maternels en relais petite enfance. Ils deviendraient ainsi de véritables lieux de référence pour les parents recherchant un mode d'accueil et des lieux ressources pour les assistants maternels,

Citons également l'introduction d'un référentiel national définissant les exigences en matière de locaux pour les établissements, opposable partout en France, pour faciliter les démarches des porteurs de projets. Enfin, le ministère des solidarités et de la santé a souhaité que cette réforme permette de refonder l'accompagnement des équipes en matière de santé du jeune enfant, afin de permettre davantage de prévention en matière de santé et d'encourager un accueil plus inclusif pour les enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques. Conformément au souhait du Parlement, la réforme favorise les expérimentations. Il est par exemple proposé d'expérimenter partout en France une obligation d'organisation de temps d'analyse de pratiques dans les établissements- demande des professionnels. De même, sera expérimenté un assouplissement des règles d'encadrement permettant qu'un seul professionnel accueille seul jusqu'à trois enfants entre dix-huit heures et six heures, afin de développer l'offre d'accueil en horaires atypiques pour les parents travaillant en horaires décalés ou ceux dont les temps de trajet nécessitent de laisser leur enfant un peu plus tôt le matin.

le coût des mineurs non accompagnés et des jeunes majeurs. Le nombre de jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) ne cesse de grimper : il a progressé de 11 % en un an- un niveau jamais atteint précédemment. Les dépenses liées à cette prise en charge se sont élevées à 15,3 millions d'euros en 2018, alors que la compensation de l'État n'a été que de 2,3 millions d'euros, soit 13 millions d'euros restant à la charge du département du Bas-Rhin.

La politique d'accompagnement des jeunes majeurs dans le département du Bas-Rhin, qui est d'ailleurs à saluer, s'appuie sur une prise en charge globale avec hébergement et accompagnement éducatif près de 6 200 enfants et jeunes sont accompagnés ou confiés à l'ASE au 31 décembre 2019 ; sur les 2 977 situations de placement, 389 sont devenus majeurs

Les nouvelles arrivées ne sont pas compensées par les sorties à 18 ans, et ces jeunes majeurs, que le département continue de prendre en charge, ne sont pas comptabilisés dans la clé de répartition. Il s'ensuit une insuffisance de l'engagement financier de l'État, lequel ne veut pas voir l'enjeu fondamental que recouvre la prise en charge de ces jeunes et laisse les départements seuls face à cette responsabilité.

accompagnés ? Faute de prise en compte des jeunes majeurs, le département doit-il renvoyer ces jeunes majeurs vers l'État et abandonner sa politique d'insertion ?

s'agissait de permettre une compensation plus juste des dépenses engagées par les départements, sur la base d'un forfait de 500 euros par jeune évalué, dont 90 euros pour la réalisation d'un examen médical obligatoire, auxquels s'ajoutent 90 euros par

conformément à l'article 51 de la loi du 10 septembre 2018, nous avons déployé un outil d'appui à l'évaluation de la minorité, le fameux fichier AEM, qui vise à faciliter et fiabiliser l'évaluation, par chaque département, de la situation des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés. Cet outil est opérationnel depuis le 7 février 2019. Nous ne l'avons pas rendu obligatoire, mais,

Aucun secteur d'activité n'est épargné, aucune zone géographique. Selon la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises), un tiers des entreprises renoncent à recruter, abandonnant du même coup des marchés supplémentaires, privant notre pays de cette croissance dont il a tant besoin. l'Essonne, que j'ai l'honneur de représenter, n'est pas épargné par cette crise de l'emploi. Tant s'en faut ! Dans leur écrasante majorité, les entreprises que je visite lors de mes nombreux déplacements sur le territoire me font part de leur forte demande de recrutement restant, malheureusement, sans résultat. C'est un énorme gâchis En même temps, le chômage, certes en légère baisse, atteint toujours 8,7 % et plus de 3,5 millions de personnes sont indemnisées par Pôle emploi. Cherchez l'erreur Inadéquation entre l'offre et la demande, déficit d'image de certains métiers, conditions de travail, niveau des salaires, les explications avancées sont multiples. La formation est sans doute une des réponses. La réforme de l'apprentissage s'inscrit précisément dans cette logique. Il en va de même pour celle de la formation, mais il est à craindre, en pratique, que le nouveau dispositif soit plus complexe. Une chose est certaine, les PME employant entre 50 et 300 salariés sont les grandes perdantes. Qu'entendez-vous faire concrètement, madame la ministre, pour corriger cette situation ? Personne ne peut plus nier, par ailleurs, qu'il faut de toute urgence établir un meilleur équilibre entre assistanat et incitation à la reprise d'un emploi. Aujourd'hui, il est possible pour un salarié à qui son employeur propose un CDI en fin de CDD de refuser et ... de s'inscrire à Pôle emploi en même temps Là encore, il faut agir ! De vraies mesures, plus fortes, plus profondes, plus pérennes, sont absolument nécessaires. Qu'entendez-vous faire concrètement, madame la ministre, pour aider nos entreprises ?

que du plan d'investissement dans les compétences, qui vise précisément à réduire l'écart entre les compétences demandées et les compétences disponibles sur le marché du travail. Après trente ans de chômage de masse, bien des compétences

Chaque emploi compte

de la justice. Madame la garde des sceaux, j'appelle votre attention sur la nécessité, pour la Chancellerie, de libérer rapidement les locaux vendus par la chambre de commerce et d'industrie de Touraine et toujours occupés par le greffe et le tribunal de commerce de Tours. Comme vous le savez, les fortes baisses de dotations budgétaires ont contraint la CCI de Touraine à mettre en vente son patrimoine immobilier. Le 4 décembre dernier, la CCI a donc vendu à un promoteur immobilier son siège situé au centre-ville de Tours. Depuis de nombreuses années, la CCI de Touraine hébergeait, à titre gratuit, le greffe et le tribunal de commerce. Le 20 décembre 2018, le ministère de la justice s'était donc engagé, par courrier, à libérer le bâtiment concerné au cours du premier semestre de 2020. En dépit de cet engagement, pourtant renouvelé au mois de septembre dernier, le greffe et le tribunal de commerce n'ont pas libéré les locaux. Plus inquiétant encore, un récent courriel adressé, semble-t-il, par le ministère à l'acquéreur fait état d'une impossibilité de libérer les locaux avant le mois de décembre 2021. Cette décision bloque le début des travaux et met en difficulté l'acquéreur, une PME régionale. Le versement d'une partie du prix de vente est évidemment conditionné à la libération des locaux. Aussi, le non-respect par le ministère de ses engagements place cette CCI, que j'ai présidée pendant plusieurs années, dans une situation financière intenable. financière intenable. Le greffe et le tribunal de commerce pourront-ils rapidement libérer les locaux vendus par la CCI, qu'ils occupent aujourd'hui sans titre et, donc, à proprement parler d'une façon illégale

qui ne permettent pas d'envisager le transfert du tribunal d'instance avant le premier semestre de 2021 et, par voie de conséquence, le déménagement du tribunal de commerce en suivant. En tout état de cause, la décision d'inutilité versée par le notaire à l'acte de vente précisait : « De façon anticipée, sont déclarés inutiles les locaux cités à l'article 1, à compter du 30 juin 2020, sous réserve de la disponibilité des locaux actuels du tribunal d'instance de Tours, après son installation au 100, rue Marceau et boulevard Béranger à Tours à l'issue d'une opération immobilière de restructuration. Ce départ ne pourra dépasser le délai légal de trois ans maximum à compter du déclassement décidé par les

pour libérer les locaux au plus tôt et, en tout état de cause, avant la date légale du 26 novembre 2021. S'agissant des éventuels préjudices financiers que vous évoquez, le vendeur ne pouvait pas ignorer les réserves portant sur la date de libération indiquée dans la déclaration d'inutilité produite dans les documents de l'acte de vente. Il doit normalement en avoir tenu compte. Enfin, la libération des locaux occupés par le tribunal de commerce et son greffe, vertu d'une ordonnance royale de 1822, s'effectuera aux frais du ministère de la justice, qui supportera bien entendu le coût du déménagement et de la prise à bail de substitution.

de notre pays depuis plusieurs années. Alors que ces entreprises apportent des solutions pour notre agriculture, qu'elles exercent leur travail de sélection et de production de semences en toute légalité, elles subissent tous les ans des destructions de parcelles de sélection ou de production de semences. Ces actes de vandalisme, perpétrés par des activistes qui se revendiquent de collectifs de citoyenneté, mais agissent sur des fondements purement idéologiques, pénalisent des activités de recherche parfaitement légales. Ils portent un coup au développement de variétés répondant aux attentes des marchés et des agriculteurs français tout en accentuant le climat de suspicion dans les territoires. L'été dernier encore, plusieurs parcelles de variétés de tournesol à forte teneur en acide oléique, recherchées précisément pour leur qualité alimentaire, et des parcelles de sélection de variétés de maïs économes en eau et en azote ont été détruites. Au-delà des pertes économiques causées aux entreprises et de la négation du travail des équipes et des agriculteurs, ces destructions peuvent retarder considérablement- jusqu'à sept ans -la mise à disposition de variétés innovantes aux agriculteurs. D'après une enquête récente menée par l'Union française des semenciers, trente-cinq destructions ont été enregistrées au cours des dix dernières années ; vingt-huit ont fait l'objet de dépôts de plainte, qui, la plupart du temps, n'ont pas été suivis d'enquête de la part de la gendarmerie seulement six procès ont été engagés, dont certains ont abouti à la relaxe pure et simple des faucheurs. Dans un certain nombre de cas, les procédures pénales sont jugées disproportionnées par rapport au préjudice subi. Il est essentiel de faire cesser la quasi-impunité des auteurs de ces destructions de cultures : à force de laxisme, on s'oriente vers une situation privant les exploitations agricoles de leur compétitivité et nos entreprises de leurs capacités de recherche. De tels actes fragilisent l'une des plus belles filières de semences

font l'objet d'une grande attention de mes services, ainsi que des procureurs généraux et des procureurs de la République, qui sont investis dans la lutte contre les atteintes commises à l'encontre des agriculteurs. À ce titre, une dépêche a été diffusée par la direction des affaires criminelles et des grâces de mon ministère le 22 février 2019 au sujet des actions violentes menées par des mouvements radicaux, et plus particulièrement par ceux qui se livrent à des intrusions sur des sites agricoles. Dans cette instruction générale, j'invite les parquets renforcer la prévention des débordements et je leur rappelle les qualifications pénales pouvant être retenues dans ces situations. Cette récente dépêche mentionne notamment que la destruction volontaire du bien d'autrui peut être retenue lorsque l'intrusion dans l'exploitation a entraîné la destruction matérielle de certains biens. L'infraction de violation de domicile permet également de répondre efficacement aux intrusions au sein des exploitations agricoles. S'agissant de la destruction de plants de semences, les différentes circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces relatives aux enquêtes, aux poursuites et à la réponse pénale applicables aux actes de destruction de ces plants invitent systématiquement les parquets à poursuivre les auteurs de tels faits avec rigueur et fermeté. Dans ce cas, on privilégie les procédures rapides, notamment la comparution immédiate. Ainsi, au mois de juin 2019, la cour d'appel de Nancy a confirmé la condamnation de cinquante-trois individus pour destruction de parcelles de culture de variétés innovantes ; quarante-neuf d'entre eux ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis. Cette réponse judiciaire atteste de la prise en compte par les parquets du trouble à l'ordre public inacceptable que provoquent ces destructions de cultures et de l'efficacité du cadre juridique actuel. j'ai rencontré récemment des parlementaires et, le 7 janvier dernier, les représentants de la FNSEA. Évidemment, j'ai été très sensible aux inquiétudes qu'ils ont manifestées. J'ai donc demandé à mon ministère que soient engagées

s'agissant des exploitations agricoles. D'autres dispositifs peuvent venir conforter ces évolutions. Cette question fera, de ma part, l'objet de nouveaux échanges avec les représentants du monde agricole et avec les parlementaires. En effet, nous devons être extrêmement attentifs et vigilants face à ces sujets.

Sur ce sujet, j'ai été rapporteur d'un certain nombre de textes. Dès 2018, à l'époque de la directive, le législateur avait proposé 75 000 euros, voire 150 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Nous en sommes bien loin ! La

Ma question porte sur l'expérimentation du contrôle des conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français. Monsieur le ministre, je sais l'attention que vous accordez à ce La multiplication de révélations de cas de maltraitance a jeté le doute sur les 263 abattoirs du pays. Il est devenu indispensable de redonner confiance aux éleveurs et aux consommateurs dans la filière d'abattage. La protection animale doit devenir pour les abattoirs un enjeu aussi important que les conditions sanitaires et les conditions de travail des salariés. Depuis plusieurs années, le Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire préconise le renforcement des contrôles et la mise en place de caméras au niveau des postes de saignée. Toutefois, l'article 71 de la loi dite « Égalim » se contente contente de prévoir la mise en oeuvre, à titre expérimental et sur la base du volontariat, pour une durée de deux ans, d'un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort. Il s'agit d'évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal. Un décret du 26 avril 2019 précise les conditions de mise en place de cette expérimentation. Les exploitants d'abattoir devaient candidater avant le 28 décembre 2019. Aussi, je souhaite savoir combien d'exploitants se sont portés candidats et les critères qui ont permis de choisir ceux qui participeront à cette expérimentation. Enfin, quel est le nombre de participants définitivement retenus et quelle est leur répartition géographique

le code minier actuel nécessite en effet une refonte totale. Aujourd'hui, les projets miniers se heurtent systématiquement à la contestation des populations en raison des risques et des larges insuffisances des procédures minières et du dispositif après-mine existants. Les bassins miniers rencontrent de nombreux problèmes, qui mettent les territoires en grande difficulté. Le dispositif après-mine doit donc être amélioré, qu'il s'agisse de l'indemnisation des dégâts ou de la gestion des risques résiduels. Le dispositif d'indemnisation actuel a ses limites il manque d'efficacité, de rapidité et d'équité. L'origine minière des dommages est souvent difficile à prouver, notamment lorsqu'ils sont liés aux terrils ou aux installations hydrauliques de sécurité. La notion de dommage minier doit donc être clarifiée. Pour les victimes les plus fragiles, il est impératif de simplifier les conditions de garantie de l'État, afin d'éviter des procédures longues qui pourraient se révéler spoliatrices. En outre, le financement de l'indemnisation doit maintenant être pris en charge par l'État sur des crédits spécifiques de l'après-mine. la gestion des risques miniers résiduels doit être améliorée à l'occasion de la future réforme, avec la mise en place d'une concertation réellement effective au niveau tant local que national. Le plan de prévention des risques miniers est un outil largement utilisé, mais avec des méthodologies différentes d'un département à l'autre. Il faut donc uniformiser cette méthodologie nationale pour que cessent les disparités de pratiques. Il est aussi nécessaire de créer une nouvelle catégorie de plan de prévention des risques propre à l'activité minière. Cette solution permettrait de gérer et de prévenir les risques miniers avec une juste indemnisation.

du code minier ainsi que les orientations du Gouvernement sur cette réforme urgente et indispensable de l'après-mine. La parole

mai 2019 et devrait être présentée en conseil des ministres au cours de l'année 2020. L'objectif est d'apporter des réponses concrètes aux parties prenantes quant à l'obsolescence des procédures minières et d'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux et socio-économiques qui concernent toute la vie des projets miniers. Cette réforme est destinée à mieux gérer et encadrer les nouveaux projets miniers. Plusieurs adaptations législatives seront donc apportées au dispositif actuel de prévention des risques miniers. Le but est d'améliorer encore la prise en compte des intérêts environnementaux. Il est par exemple envisagé d'ajouter la prise en compte des risques sanitaires dans le code minier. Il est aussi prévu d'inclure les travaux miniers dans l'autorisation environnementale, ce qui permettra de mettre en cohérence les procédures d'instruction au sein du code de l'environnement et de bénéficier de dispositions harmonisées concernant les contrôles et sanctions administratifs. Il est également envisagé d'étendre les garanties financières pour les travaux d'exploitation miniers à la remise en état du site après fermeture. Ces mesures nouvelles compléteront les moyens importants que l'État pour assumer sa responsabilité en matière d'après-mine. Ainsi, mon ministère consacre chaque année près de 40 millions d'euros de crédits spécifiques à la réparation des dommages miniers et à la prévention des risques en Je précise que la garantie apportée par l'État dans la réparation des dommages miniers n'est valable qu'en cas de disparition ou de défaillance du responsable minier. Pour autant, dès lors que cette condition est vérifiée, la prise en charge par l'État peut avoir lieu, qu'il y ait ou non un plan de prévention des risques miniers sur le territoire concerné. La

la ministre de la transition écologique et solidaire. Lors du sommet franco-italien du 27 septembre 2018, le Président de la République a confirmé l'engagement de notre pays dans la réalisation du tunnel international du Lyon-Turin. Nous nous félicitons des étapes franchies et de l'inauguration des neuf premiers kilomètres déjà réalisés, en vue d'une mise en service en 2030 de la section transfrontalière. L'autre étape importante annoncée par la coordinatrice européenne est le fait que la Commission européenne du financement, sa participation à 55 % pour le tunnel de base et à 50 % pour les accès depuis la métropole lyonnaise. L'enjeu est donc aujourd'hui d'ouvrir rapidement ce deuxième volet. Le 8 avril 2019, le Gouvernement a engagé un programme d'études pour préciser les investissements nécessaires et le phasage possible. Pour rester dans un calendrier cohérent, le Parlement a inscrit dans la loi d'orientation des mobilités l'échéance de 2023. Or la Commission européenne vient de lancer un appel à projets au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, les dossiers devant être déposés avant le 28 février 2020 : la date limite porte sur 500 millions d'euros de subventions communautaires, auxquelles seraient éligibles les études de phasage des voies d'accès. Lors du sommet franco-italien qui s'est tenu à Naples il y a quelques jours, les deux gouvernements ont décidé d'entamer « au niveau politique, un " dialogue stratégique sur les transports " pour définir, entre autres, la demande et les conditions de financement européen des voies d'accès au tunnel de base, ainsi que le soutien à l'autoroute ferroviaire alpine ». Or, concernant cette autoroute, un appel d'offres a été lancé il y a maintenant dix ans pour une délégation de service public, et nous attendons toujours la décision du Gouvernement. Concernant les accès, l'Europe, qui a fait savoir sa disponibilité pour un financement à 50 %, attendait également d'être sollicitée pour l'appel d'offres arrivé à échéance il y a quelques jours.

Lyon-Turin, et cet engagement a été repris dans la LOM, promulguée le 26 décembre 2019. Ce projet est en effet stratégique pour améliorer l'environnement des vallées alpines et sécuriser les flux de transports entre la France et l'Italie, lesquels reposent aujourd'hui presque exclusivement sur des passages routiers.

à court terme du réseau existant et de préciser la consistance et le phasage des lignes nouvelles des accès français. La LOM fixe à 2023 l'échéance pour solliciter un cofinancement européen au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Le Gouvernement n'a pas attendu cette échéance pour prendre ses responsabilités : je vous confirme que, dans le cadre de l'appel à projets européen dit « reflow call », nous avons déposé un dossier visant à bénéficier de subventions européennes. Celui-ci porte sur les 4 millions d'euros de dépenses éligibles, pour un cofinancement européen attendu jusqu'à 50 %. Les résultats de cet appel sont prévus pour juillet. Une fois cette démarche aboutie, la consistance et le calendrier des opérations clairement définis, soyez assuré que nous veillerons à solliciter de nouveau les financements associés. Le prochain mécanisme pour l'interconnexion en Europe pour la période 2021-2027 sera probablement un des vecteurs majeurs pour subventionner, au niveau européen, des études plus abouties sur ces accès. Soyez ainsi assuré, monsieur le sénateur, de notre pleine volonté d'agir pour ce projet d'ampleur nationale et européenne sur lequel nous vous savons très mobilisé,

le champ de leurs missions en couvrant désormais une population près de cinq fois supérieure. Dans le même temps, la filière nucléaire doit toujours faire face à des défis multiples : poursuite de l'exploitation d'installations vieillissantes, construction de nouvelles infrastructures de type EPR ou encore débat public engagé sur la gestion des déchets liés à l'activité nucléaire. Les moyens financiers alloués par l'État, l'Autorité de sûreté nucléaire, n'ont pourtant connu qu'une réévaluation très modeste ces dernières années. L'an passé, les CLI ne disposaient plus pour oeuvrer, du fait de l'extension de leur périmètre d'intervention, que de 22 centimes par habitant, contre encore 87 centimes en 2018. Pour garantir leur fonctionnement efficient, il conviendrait que que l'État maintienne au moins, au bénéfice des CLI et de l'Anccli, un niveau de ressources par habitant équivalent à celui qui était en vigueur avant l'élargissement de leur périmètre d'intervention. Pour ce faire, un budget d'environ 5 millions d'euros serait nécessaire. La loi relative à la transparence et à la sécurité nucléaire de 2006 a prévu d'attribuer une partie de la taxe sur les installations nucléaires de base à leur fonctionnement, mais, jusqu'à maintenant, elles n'ont pas pu en bénéficier.

et je ne peux que défendre la pertinence d'une telle implication de la société civile dans la question nucléaire dans notre pays. Nous savons, en effet, que la culture du risque en matière nucléaire n'est pas parfaitement assimilée en France et que les réflexes requis en cas d'incident sont encore largement méconnus de la population. La distribution des pastilles d'iode entreprise depuis plusieurs mois dans la nouvelle bande des dix à vingt kilomètres n'a d'ailleurs, à ce jour, trouvé écho en moyenne qu'auprès d'un cinquième de la population concernée et d'une proportion plus faible encore des établissements accueillant du public. Madame la secrétaire d'État, compte tenu de ces enjeux, le Gouvernement envisage-t-il une revalorisation significative des moyens des CLI et de l'Anccli dans le cadre de l'élargissement de leurs missions ? ? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice, vous appelez notre attention sur la situation financière des CLI dans le contexte de l'extension du périmètre des plans particuliers d'intervention des centrales nucléaires de production d'électricité.

les missions qui leur ont été confiées par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. En France, une commission locale d'information est mise en place pour chaque installation nucléaire. Les CLI rassemblent des représentants de la société civile et constituent à la fois des interlocuteurs incontournables des exploitants et des autorités. Elles ont donc une double mission informer la population sur les activités nucléaires et assurer un suivi permanent de l'impact des installations nucléaires. Leur activité n'est donc pas proportionnelle à la population qui figure dans le périmètre des PPI. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, sur mon initiative, a sollicité Parlement pour obtenir une augmentation des ressources budgétaires des CLI à hauteur de 1,3 million d'euros. Dans le contexte actuel de modération budgétaire, il s'agit d'un effort important, auquel auquel s'ajoutent les moyens récemment mis en place en faveur de la transparence et de l'information sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Enfin, le mécanisme d'affectation budgétaire que vous rappelez ne pourrait s'appliquer

établis conformément au cadrage national. Ils répondent à deux priorités du Gouvernement : un recentrage des interventions dans une logique de solidarité territoriale, principalement envers les territoires ruraux, ainsi que la poursuite et le renforcement des interventions en faveur de la préservation des milieux aquatiques, de la biodiversité et des milieux marins. Concernant l'eau potable et l'assainissement, les agences de l'eau accompagnent financièrement des collectivités qui sont en difficulté structurelle parce qu'elles sont situées en zones de faible densité de population et de faible potentiel fiscal et pour lesquelles un juste prix de l'eau ne permet pas de faire face aux besoins d'investissement ou de renouvellement de leurs équipements. La question plus spécifique de l'aide à l'assainissement non collectif a largement été débattue lors des discussions portant sur les onzièmes programmes. En raison d'enjeux environnementaux généralement faibles et dans l'objectif de davantage les interventions des agences de l'eau, qui concourent à la reconquête de la qualité des eaux et à la préservation de la biodiversité, l'assainissement non collectif n'a pas été retenu parmi les priorités ministérielles. Les comités de bassin étaient ainsi invités à les décliner au mieux en fonction de leurs enjeux propres. Certains d'entre eux ont fait le choix de ne pas totalement abandonner les aides en faveur de l'assainissement non collectif, mais de les limiter. Ces solutions, issues de discussions qui se sont tenues au sein des comités eux-mêmes, m'apparaissent comme un compromis pragmatique, dans la mesure où elles contribuent pleinement à l'amélioration de la qualité des masses d'eau. les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation ou de réhabilitation de leurs installations d'assainissement non collectif peuvent bénéficier d'autres dispositifs d'aides,

Depuis plus de vingt ans, la mise à deux fois deux voies de la route nationale 19, qui va de Langres à la Suisse, progresse trop lentement, au rythme imposé par le niveau limité des enveloppes budgétaires successives mobilisées par l'État. La RN 19 est pourtant une route dont l'État a souhaité conserver la propriété au regard de ses enjeux structurants en termes d'aménagement et de développement du territoire. Si les dispositions du contrat spécifique à la RN 19 ont été scrupuleusement respectées par tous les gouvernements, notamment la clé de financement des travaux fixée à hauteur de 75 % pour la part de l'État et à 25 % pour celle des collectivités locales, la Haute-Saône n'a, à ce jour, plus de visibilité à long terme sur l'avenir de cet axe. La seule information officielle concerne le tronçon ouest, entre Port-sur-Saône et Langres, dont le nouveau parti d'aménagement annoncé en 2019 par la ministre des transports ne prévoit plus que des travaux ponctuels, tels que des contournements de villages ou des sécurisations de carrefours, ce qui est inadmissible. C'est pourquoi je souhaite savoir si la mise à deux fois deux voies de la totalité du tronçon entre Amblans et Vesoul reste une priorité pour l'État et si la clé de financement des travaux restera conforme dans le contrat spécifique à la RN 19. Je souhaite, enfin, connaître le délai de la négociation sur la priorisation et sur le montage financier des prochains

! La parole est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, l'aménagement de la RN 19 entre Vesoul et Amblans-et-Velotte fait partie d'un programme de mise à deux fois deux voies entre Vesoul et Lure, déclaré d'utilité publique en 2005. La réalisation d'une première section entre Amblans-et-Velotte et Lure a été inscrite au CPER 2015-2020 de la région Bourgogne-Franche-Comté et a été mise en service en 2017. Cet aménagement représente un investissement important, financé à 75

Comme l'a rappelé Élisabeth Borne en juillet dernier en réponse à la sollicitation de M. Houlley, maire de Lure, l'État reste pleinement mobilisé dans l'aménagement à deux fois deux voies de la section restante de la RN 19 entre Vesoul et Amblans-et-Velotte. C'est pourquoi, malgré l'absence de ligne de financement spécifique dans le CPER actuel, il mène les études de conception détaillée du projet et a acquis le foncier nécessaire la réalisation de la deux fois deux voies dans cette dernière section. Les travaux de cette opération ne pourront cependant être réalisés que dans le cadre d'une prochaine contractualisation entre l'État et la région, qui viendra, en particulier, définir les modalités de leur financement. L'État investit déjà massivement en Haute-Saône, notamment dans le cadre du CPER actuel, au travers du projet de déviation de Port-sur-Saône sur la qui représente un investissement de plus de 130 millions d'euros, dont plus de 97 millions d'euros apportés par l'État. Tout en confirmant la volonté de l'État de mener à terme la mise à deux fois deux voies de la RN 19 entre Vesoul et Amblans-et-Velotte, je vous précise qu'une implication forte des collectivités dans le financement de ce projet ne pourra qu'accélérer

dès cette année d'échanges avec les régions, en parallèle à la négociation des nouveaux CPER. L'enveloppe budgétaire pour la région Bourgogne-Franche-Comté n'est donc pas encore connue à ce jour. Merci de votre présence,

La présidence du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) est vacante depuis le 31 octobre 2019. Au moins cinq personnalités ont présenté leur candidature pour ce poste,

Selon les informations de la presse, confirmées par l'intéressé, M. Thierry Coulhon, conseiller à la présidence de la République, aurait fait acte de candidature.

permettez-moi de profiter de votre question pour rendre hommage à l'immense travail réalisé par le HCERES sous la présidence de Michel Cosnard depuis 2015, qui laissera une empreinte durable que nous tâcherons de faire vivre à l'avenir. faire vivre à l'avenir. La nomination du président du collège du HCERES est une compétence du Président de la République en conseil des ministres, conformément à la loi organique visant à préciser les dispositions de l'article 13 de la Constitution. Un appel à candidatures a été ouvert par mon ministère afin de préparer cette nomination, laquelle ne pourra intervenir qu'après consultation des commissions permanentes compétentes des deux assemblées. Vous serez donc informé dans les meilleurs délais du nom de celui ou de celle qui sera proposé à ces fonctions, selon les procédures d'ores et déjà prévues par les textes. Vous l'avez mentionné, parmi les différents dossiers adressés au ministère, une candidature collective a été présentée par plusieurs centaines de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. J'en profite pour remercier les services du ministère qui ont instruit ces candidatures.

précise les attributions et les compétences du président du collège, désigné comme étant une personne nommée par décret en conseil des ministres. C'est le collège du HCERES qui est le lieu de la collégialité, non sa présidence, qui n'est pas une fonction collective. Dans ces conditions, un collège de plusieurs centaines d'enseignants-chercheurs ne pouvait donc être assimilé à une seule et même personne. Ensuite, cette candidature multiple était avant tout un moyen de faire connaître un certain nombre d'interrogations, voire de craintes, contenu du projet de loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, qui sera bientôt finalisé. Les directeurs généraux de mon ministère ont tâché de transmettre par courrier une première série de réponses aux inquiétudes exprimées, notamment sur la question des revalorisations indemnitaires qui interviendront dès l'année prochaine. J'aurai naturellement l'occasion de m'exprimer plus largement sur ce sujet, comme j'ai pu le faire auprès de la communauté académique. Nous aurons, de plus, un débat en séance publique, puisque votre groupe a demandé l'inscription le 24 mars prochain d'un débat sur la politique de recherche publique en France, auquel je participerai évidemment avec un grand plaisir. Merci

Les maires de ces petites communes sont très investis sur cette question et se battent quotidiennement pour améliorer la situation afin de répondre à une demande légitime des habitants et des entreprises. La complexité et la lenteur des procédures ne sont pas acceptables. Après avoir effectué, parfois à plusieurs reprises, des mesures prouvant l'absence de réseau de téléphonie mobile sur un territoire, il faut attendre l'arrêté attestant la reconnaissance de l'existence d'une zone blanche. C'est une première étape, mais l'obtention de cette reconnaissance n'est pas synonyme d'une résolution rapide du problème, et de nouveaux délais s'imposent aux élus locaux. Même lorsque les antennes-relais sont montées, il faut parfois attendre plusieurs mois avant qu'elles ne soient connectées au réseau de téléphonie mobile. L'incompréhension L'incompréhension des élus face à ces retards est par ailleurs accentuée par la multiplicité des interlocuteurs auxquels ils ont affaire lorsqu'ils essaient d'obtenir des réponses claires auprès des opérateurs. exemple parmi d'autres : la commune de Saint-Paul-du-Bois est actuellement confrontée à ces difficultés depuis plusieurs années. Après plusieurs séries de mesures effectuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), cette commune a été reconnue zone blanche prioritaire. Malgré cette reconnaissance- elle-même tardive -, d'importants délais ont été annoncés aux élus locaux avant la mise en place effective d'une antenne-relais. Ce cas n'est pas isolé plusieurs communes se trouvent dans des situations similaires. Monsieur le ministre, compte tenu des enjeux importants que revêt une couverture mobile de qualité en termes d'attractivité et de développement du territoire notamment, quelles mesures comptez-vous prendre pour faciliter et accélérer la mise en place effective des antennes-relais dans les territoires

Depuis la signature de cet accord en janvier 2018, plus de 5 000 communes sont passées des anciennes technologies, de la 2G ou de la 3G, aux nouvelles technologies telles que la 4G. Plus de 1 300 communes

opérateurs, on a réglé le sujet. J'invite donc vos interlocuteurs à se rapprocher de l'équipe projet de Maine-et-Loire. Enfin, sur la question de l'interlocuteur unique à ces équipes projets, nous avons créé, au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, un dispositif, l'Agence France mobile,

une forme de légèreté d'application de la loi SRU serait catastrophique pour la production de logement social dans notre pays.

Le 26 septembre dernier, les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime ont été engagés pour lutter contre un violent incendie de l'usine Lubrizol, entreprise classée « Seveso, seuil haut », à Rouen. Ce sinistre d'intensité exceptionnelle a produit un important panache de fumée, qui a conduit le préfet à déclencher le plan particulier d'intervention du secteur concerné en vue d'assurer la protection des populations. À cette occasion, la conjonction des moyens du SDIS de la Seine-Maritime, de ceux d'autres SDIS et de moyens privés engagés en renfort a permis d'éteindre l'incendie en moins de douze heures sans faire de victime, ni parmi les personnes engagées ni dans la population. ce sinistre est considérable en termes de moyens humains et matériels. À l'évidence, les ressources actuelles du SDIS de la Seine-Maritime ne lui permettent pas de faire face, à lui seul, à un accident industriel majeur de l'ampleur de celui de l'usine Lubrizol, que l'on peut qualifier de hors norme, tant il a dépassé les enveloppes habituellement retenues pour ce type de dangers. Plus largement, la défense des quelque soixante-sept sites « Seveso » de la Seine-Maritime pose aujourd'hui clairement la question du dimensionnement de notre réponse capacitaire en matière de couverture des risques dits particuliers. Sans l'intervention de très grande qualité des sapeurs-pompiers, l'incendie de l'usine Lubrizol aurait eu des répercussions autrement plus catastrophiques pour la métropole de Rouen. Il est donc nécessaire de tirer rapidement tous les enseignements de ce sinistre, sans occulter la question des coûts supportés par les SDIS pour ce type d'opérations. Aussi je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir préciser

de la réponse capacitaire des SDIS face à des risques particuliers, le ministre de l'intérieur a annoncé, le 21 octobre dernier, la mise en place dans chaque département d'un pacte capacitaire. Cette démarche doit permettre d'offrir une visibilité pluriannuelle sur les investissements et les budgets de ces services. La construction de ces pactes consistera à organiser la mise en commun, à l'échelle de la zone de défense et de sécurité, des éléments mis en évidence par les différents schémas départementaux d'analyse et de couverture

on le sait, ils connaissent de très sérieuses tensions budgétaires, qui limitent leur capacité à investir pour faire face aux risques particuliers, notamment aux risques industriels majeurs.

soulignant la dégradation rapide du vivre ensemble, les actes délictueux et les incivilités au quotidien qui s'accroissent, exacerbant les tensions sociales.

de Castillon-la-Bataille, qui a appelé mon attention sur la situation spécifique de sa commune. Par un courrier du 15 novembre dernier, il a relayé auprès de vos services ses inquiétudes relatives à l'absence de renforts de gendarmerie mobile affectés

la voie publique et aménagé un logement pour loger les effectifs supplémentaires de gendarmerie annoncés. Toutefois, depuis un an, une hausse des atteintes aux personnes et aux biens est à déplorer.

Ensuite, le groupement de gendarmerie départementale de la Gironde a pris des mesures opérationnelles visant à renforcer la présence des gendarmes départementaux pour rassurer la population et prévenir les incivilités. Enfin, des services de surveillance réalisés par des réservistes opérationnels sont quotidiennement programmés au profit de la communauté de brigades de Castillon-la-Bataille. Ces efforts importants ont vocation à s'inscrire dans la durée.

J'appelle l'attention du Gouvernement sur le renouvellement des concessions hydroélectriques de la vallée de la Têt, dans les Pyrénées-Orientales. L'hydroélectricité est la première énergie renouvelable en France. Flexible, elle contribue fortement à la transition énergétique, un enjeu majeur. Or la filière hydroélectrique est aujourd'hui dans l'expectative. En effet, la question du renouvellement des concessions hydroélectriques, ouverte depuis maintenant plus de dix ans, a connu plusieurs rebondissements une mise en concurrence annoncée en 2012, une mission parlementaire, puis des modalités intégrées dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sans oublier deux mises en demeure de la Commission européenne. elle a été évoquée lors des réflexions sur la réorganisation d'EDF ; dans le cadre du projet Hercule, il s'agirait de regrouper les concessions hydroélectriques de cet opérateur dans une entité nationalisée. Toutefois, ces réflexions semblent ajournées, dans l'attente des discussions avec l'Europe sur l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique.

Cette piste est en cours d'étude, après avoir fait l'objet de premiers échanges avec la Commission européenne. À ce stade, aucune décision n'a été prise. Le renouvellement des concessions, par remise en concurrence ou une structure 100 % publique, est une politique nationale que nous souhaitons mener en vue d'optimiser la gestion des barrages et de relancer l'investissement dans ce domaine, tout en redistribuant des ressources financières vers les territoires. Par ailleurs, une attention particulière sera évidemment portée aux personnels des sociétés exploitantes. Quelle que soit la solution retenue pour la gestion des concessions hydroélectriques, soyez certain que nous accorderons une attention spéciale aux grands opérateurs et à leur potentiel énergétique, technique et humain, mais aussi aux concessions qu'ils exploitent. La parole est

Las, le 24 décembre 1986, la mine a fermé, victime d'un effondrement des cours du tungstène orchestré par la Chine. La Chine qui, aujourd'hui, a le monopole de l'extraction et de la mise sur le marché de ce matériau rare, qui constitue un des éléments de fabrication essentiels pour les objets des nouvelles technologies. Si la mine de Salau renfermait encore un gisement important de tungstène, cela constituerait un enjeu stratégique pour l'économie française, plus particulièrement pour l'économie ariégeoise. En novembre 2014, la société Variscan demande de permis exclusif de recherche minière, accordé le 21 octobre 2016 par le secrétaire d'État chargé de l'industrie. Toutefois, le 28 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis pour vice de forme. Très rapidement, le ministère de l'économie a fait appel de cette décision et demandé le sursis à exécution du jugement. Dernier rebondissement en date : le 24 octobre dernier, la société Variscan Mines, qui soutenait le projet de recherche minière, a demandé sa liquidation judiciaire. Compte tenu du contexte économique national et mondial, bousculé aujourd'hui par la crise sanitaire du coronavirus, la reprise des recherches sur le site de la mine de tungstène de Salau permettrait de connaître l'exact potentiel de cette zone minière, mais aussi de mesurer les risques éventuels pour l'environnement. Les riverains,

Bruno Le Maire. L'exploration minière est l'étape préalable à tout projet d'exploitation ; sans elle, il est impossible de mettre en évidence l'existence d'un gisement exploitable, sur les plans tant technique et économique que de la préservation de l'environnement.

est de classe mondiale. La faisabilité de son exploitation reste à évaluer. Cette opération doit être menée par les opérateurs miniers, qui disposent des connaissances, des compétences et des moyens nécessaires pour évaluer le potentiel du gisement et affiner les paramètres technico-économiques qui permettront le développement et le dimensionnement d'un projet minier et métallurgique pertinent sur les plans environnemental, économique et social.

Vous avez rappelé l'importance stratégique du tungstène pour notre industrie et les risques d'approvisionnement pesant sur cette ressource du fait de la position monopolistique chinoise. Le Gouvernement est pleinement conscient de ces enjeux. le Premier ministre a mis en place un groupe de travail de haut niveau, sous l'égide du Conseil national de l'industrie, afin d'élaborer un plan d'action sur la sécurisation de nos approvisionnements en métaux critiques pour les batteries, les énergies renouvelables et les alliages spéciaux utilisés par l'aéronautique et la défense. Le tungstène entrant dans la composition de ces derniers, l'ensemble des exploitations, dont celle que vous avez mentionnée, feront partie de la discussion. Pour le ministère de l'économie et des finances, il demeure essentiel que la France n'obère pas sa capacité à exploiter les ressources de son propre sous-sol, afin de réduire sa dépendance et de consolider le tissu industriel national consommateur de tungstène. Nous souhaitons aussi définir clairement une politique nationale des ressources et des usages du sous-sol, en accord avec la stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources. La parole est à M. Alain Duran,

confié la mission du service universel de téléphonie, ne parvient pas à remettre en état un réseau déjà très défectueux. La situation a encore été aggravée en 2019 par des conditions météorologiques exceptionnelles. Ainsi, certains Drômois n'avaient toujours pas accès au service téléphonique près de trois mois après les intempéries ! Ce qui signifie qu'ils n'avaient plus accès non

qui doivent remplir toutes leurs déclarations en ligne, pour des commerçants qui ne peuvent plus accepter les paiements par carte bancaire ou pour des particuliers malades ou âgés qui doivent pouvoir joindre à tout moment leur famille ou les services sanitaires et sociaux. Même si la situation s'est un peu améliorée aujourd'hui, l'état global du service de téléphonie fixe dans la Drôme est catastrophique. La devient exaspérante ! D'autant que, face aux réclamations, Orange n'apporte aucune réponse satisfaisante, semblant simplement vouloir gagner un peu de temps jusqu'au déploiement total de la fibre optique par le syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique- à nos frais plutôt qu'aux siens ... Les élus n'en peuvent plus de devoir sans cesse solliciter les services d'Orange pour des dysfonctionnements dans leur commune et, parfois, d'être mis en cause par leurs concitoyens, excédés de ne pas pouvoir accéder à des services pour lesquels les urbains ne rencontrent quasiment pas de difficultés. Pour les ruraux, cette situation contribue à renforcer leur impression de délaissement, l'impression de compter pour quantité négligeable. Le service public, le service universel, même s'il est délégué à une entreprise privée, marque la présence de l'État : il doit assurer l'égalité d'accès de tous

aggravées par les intempéries qui ont récemment frappé votre département. Le Gouvernement attache la plus grande importance à ce que tout soit mis en oeuvre pour que, à la suite de tels événements, les citoyens puissent accéder aux services essentiels auxquels ils ont droit, tels l'eau, le gaz, l'électricité et les communications électroniques, et ce dans les meilleurs délais. Le ministre de l'économie et des finances a transmis à ses services les indications dont vous nous avez fait part en ce qui concerne les difficultés rencontrées par certains citoyens pour accéder aux services de communications électroniques, notamment à la suite des intempéries dont nous avons parlé. Bruno Le Maire a mandaté la direction générale des entreprises et le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère pour organiser au plus vite une réunion avec les opérateurs de communications électroniques, notamment celui dont vous avez cité le nom, et la préfecture de la Drôme, d'établir un retour d'expérience sur cet événement et sur la manière dont ses conséquences ont été traitées, en vue d'améliorer au plus vite la situation. Nous porterons une attention particulière aux résultats de cette réunion et veillerons à ce que le cadre juridique applicable en matière de résilience des réseaux de communications électroniques soit bien respecté par tous.

ministre de l'économie et des finances. Ma question concerne l'application de la taxe d'habitation aux locaux des associations à but non lucratif. J'ai été récemment informé par le maire d'une commune du Haut-Rhin qu'une association locale de jeu de quilles s'est vu assujettir, pour la première fois en trente années d'existence, à la taxe d'habitation au titre de 2019, année où les deux tiers des ménages ne payaient déjà plus la taxe d'habitation. Interrogée, l'administration fiscale a répondu que les locaux de l'association de quilles répondaient aux conditions énumérées au 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, à savoir être « meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif », et ne pas être soumis à la taxe professionnelle. Or l'intention du Gouvernement est bien de faire disparaître progressivement la taxe d'habitation pour la totalité des foyers, quel que soit l'état de fortune des résidents. Ainsi, la loi de finances pour 2018 a initié le mouvement en prévoyant que 80 % des contribuables bénéficieront d'un dégrèvement progressif sur trois ans de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à raison de 30 % en 2018, de 65 % en 2019 et de 80 % en 2020. outre, la loi de finances pour 2020 a acté la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales à compter de 2023, au terme d'une nouvelle période transitoire pour les 20 % des foyers les plus aisés. aisés. À ma connaissance, la taxe d'habitation sur les locaux associatifs n'est pas concernée. Par conséquent, je voudrais faire remarquer qu'en 2023 la situation sera pour le moins paradoxale plus aucune résidence principale ne sera assujettie à la taxe d'habitation, quel que soit l'état de fortune de l'occupant, tandis que les locaux des associations y resteront assujettis, au même titre que les résidences secondaires.

préjudiciable à la vie associative en modifiant le 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts afin d'exempter de la taxe d'habitation tous les locaux des associations à but non lucratif. Si tel est le cas, quel est le délai envisagé ? Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie par avance de votre réponse, que j'espère positive, au nom de tous les bénévoles qui font vivre le lien social à travers ces associations à but non lucratif.

En contrepartie, elles ne contribuent pas à la cotisation foncière des entreprises. Le droit fiscal, je vous le confirme, n'a pas évolué sur ce point. Conformément à l'engagement du Président de la République, le Gouvernement a engagé un allégement de la pression fiscale pour l'ensemble des ménages, visant à augmenter le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Dans la lignée de l'article 5 de la loi de finances pour 2018, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive, par étapes, de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale. La taxe d'habitation afférente aux résidences secondaires ainsi qu'aux autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est donc maintenue. Sans Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à l'action des organismes que vous avez cités, il n'est pas envisagé, à ce stade, d'étendre la suppression de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, destinée à soutenir le pouvoir d'achat, aux autres contribuables, dont les associations sans sans but lucratif. Dans le cas contraire, ces contribuables seraient exclus de toute participation au financement des dépenses locales. En effet, cela conduirait à reporter la perte de ressources pour les collectivités territoriales sur les autres contribuables locaux, dont les ménages. Les associations éprouvant de réelles difficultés pour acquitter leur cotisation de taxe d'habitation peuvent, je le rappelle, solliciter auprès du service des impôts la remise gracieuse de tout ou partie de leurs impositions. Pour ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à la mesure que vous évoquez.

Monsieur le secrétaire d'État, j'appelle votre attention sur les conséquences de la modification du périmètre des bénéficiaires de la prime dite « Macron ». La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place l'année dernière. Cette prime, je le rappelle, est exonérée de cotisations et de contributions sociales dans la limite de 1 000 euros pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur du SMIC. Elle est également exonérée d'impôt sur le revenu dans la même limite. Cette exonération repose néanmoins sur une condition : l'entreprise devra être couverte par un accord d'intéressement ou alors en conclure un pour une durée de trois ans. Une exception existe toutefois pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique, qui sont dispensées de conclure un accord d'intéressement. Si, initialement, les députés avaient accordé cette dispense aux associations loi 1901, la rédaction finale exclut celles qui ne sont pas reconnues d'utilité publique.

Les établissements et services d'aide par le travail (ÉSAT) sont généralement des associations privées à but non lucratif. Aussi, les salariés en situation de handicap travaillant en ÉSAT se trouvent ainsi injustement pénalisés.

l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, mais dans l'objectif de développer l'intéressement, en s'appuyant sur les outils mis en place dans le cadre de la loi Pacte. C'est par un amendement parlementaire qu'il a été proposé de dispenser de la condition de conclure un accord d'intéressement certaines associations, à condition qu'elles soient reconnues d'utilité publique. Je rappelle par ailleurs que les associations peuvent tout à fait mettre en place des accords d'intéressement. En outre, la loi prévoit bien que les établissements et services d'aide par le travail sont éligibles au dispositif dans des conditions très favorables également. En effet, l'article 7 prévoit que l'exonération est applicable « aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code ». Les conditions pour que ces établissements bénéficient de l'exonération sont mentionnées plus loin : « Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II »- c'est-à-dire sous réserve des conditions de revenus, de modulation et d'égalité de traitement prévues pour l'ensemble des primes -« et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail [ ...] par un contrat de soutien et d'aide par le travail [ ...], à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V. » Il n'y a donc aucune discrimination dans l'accès au dispositif pour ces associations, qui sont au contraire favorisées puisqu'aucune condition de mise en place d'un intéressement plus pérenne n'est requise pour elle.

des comptes publics. Ma question s'adresse au ministre de l'action et des comptes publics et porte sur l'inquiétante dégradation des conditions de travail des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP ) et ses conséquences pour l'exercice de leur mission.

Ajoutons à cela la complexification de la charge de travail des agents liée à l'adoption chaque année de nouvelles dispositions fiscales. La formation des agents a également été victime de la rigueur, car la formation initiale s'est affaiblie, alors que la formation continue, elle, ne s'est pas renforcée. Mais les causes du mal-être au travail ne procèdent pas seulement du chassé-croisé entre la baisse des moyens et la hausse de la charge de travail ; elle se trouve également dans la réorientation des missions des agents. Le résultat, c'est que le mal-être au travail des agents de la DGFiP s'accroît. Outre les nombreuses remontées des services dont disposent les organisations syndicales, les différents outils mis en place par les pouvoirs publics eux-mêmes ces dix dernières années confirment cette évolution les situations de souffrance auprès des médecins de prévention au travail ont augmenté de 24 % entre 2011 et 2018. Ce résultat, on peut le penser, est sous-dimensionné par rapport à la réalité nombreux sont les fonctionnaires qui ne déclarent pas leurs souffrances. Ma question est donc la suivante : comment comptez-vous mettre fin à cette inquiétante dégradation des conditions de travail des agents et, par conséquent, améliorer l'exercice de leur mission et, partant, la qualité du service public ?

destinée à renforcer la qualité du service rendu à nos concitoyens, à diversifier les compétences de ses agents et à contribuer à une meilleure présence des services sur le territoire. Il n'est pas anormal que, dans une telle phase, des interrogations, voire des inquiétudes s'expriment. La DGFiP doit en tenir compte et y répondre. C'est pourquoi elle mène de nombreuses actions dans ce cadre. Tout d'abord, elle est à l'écoute de ses agents, avec une gamme importante d'outils leur permettant de s'exprimer sur leur travail et leurs difficultés. Cette écoute prend notamment la forme d'un dialogue social particulièrement nourri : plus d'une centaine de rendez-vous ont ainsi été proposés aux organisations syndicales de la DGFiP en 2019. Gérald Darmanin et Olivier Dussopt les ont d'ailleurs personnellement rencontrées. La DGFiP travaille également à renforcer la qualité de vie au travail. Ainsi, en 2018, elle a consacré 9,31 % de sa masse salariale à l'effort de formation, soit une progression de plus de 1 point par rapport à 2017. Chaque agent de la DGFiP bénéficie en moyenne de 4,71 jours de formation chaque année. La formation continue est donc plus que jamais une priorité pour la DGFiP, qui a engagé un ambitieux plan de modernisation visant à permettre à chaque agent d'être acteur de son parcours de formation et à faciliter les évolutions professionnelles et l'acquisition de nouvelles compétences. Par ailleurs, elle accorde une attention particulière à l'amélioration du travail au quotidien en s'appuyant sur la recherche de simplifications dans les procédures et dans l'organisation afin d'alléger la charge de travail. Celle-ci est facilitée par les outils numériques, qui permettent d'automatiser de nombreuses procédures et de recentrer ainsi l'activité des agents sur des compétences expertes. Les conditions de vie au travail, ce sont également les applications informatiques utilisées quotidiennement par les agents. Pour soutenir ces actions, en 2020, les crédits informatiques ont augmenté de 40 % par rapport à 2019, avec l'objectif de lutter contre l'obsolescence, les ralentissements et les dysfonctionnements de ces outils. La mise en oeuvre des nouveaux modes d'organisation du travail doit également permettre d'améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée des agents. Dès la première année de déploiement, en 2018, plus de 4 500 agents ont ainsi bénéficié du télétravail. Des moyens financiers importants- 7 millions d'euros -ont été consacrés à l'action sociale au profit des agents de la DGFiP et sont également mobilisés afin d'offrir des prestations sur l'ensemble du territoire. Enfin, la mise en oeuvre du nouveau réseau de proximité des ressources humaines fait l'objet d'un accompagnement personnalisé des agents concernés. Chaque agent peut ainsi bénéficier d'un accompagnement non seulement d'un point de vue financier, mais aussi pour évoluer dans ses fonctions un parcours de formation adapté en cas de changement de métier. La qualité du service rendu par la DGFiP est extrêmement appréciée, comme le démontrent toutes les enquêtes d'opinion- plus de 80 % d'approbation de son action. C'est le résultat de l'investissement des agents et des réussites collectives- comme sur le prélèvement à la source. Cet engagement reflète le fait que tous les agents de la maison ont un avenir formidable en son sein. Monsieur le

France Télécom, où le harcèlement institutionnel a été reconnu par le juge, je pense que l'État devrait globalement se poser la question des conditions de travail et des risques auxquels sont soumis les agents de la fonction publique. On observe un nombre de suicides élevé

de la jeunesse. Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur la répartition du fonds pour le développement de la vie associative. Placé sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, ce fonds a pour objet de contribuer au développement des associations. Créé par un décret du 30 décembre 2011, il a revêtu une importance grandissante depuis la suppression de la réserve parlementaire, dont une partie lui a été réaffectée. En effet, sa mission est de venir en complément de la dotation de soutien à l'investissement local, de favoriser le développement d'initiatives locales au moyen d'une enveloppe de 33 millions d'euros. Du temps de la réserve parlementaire, les élus disposaient d'une connaissance très fine de leur territoire, laquelle leur permettait de respecter une certaine équité territoriale dans la répartition des 50 millions d'euros dont ils avaient la charge et une attention particulière était accordée aux associations, y compris les plus petites, portant des projets dans les territoires les plus reculés. Alertée par un élu siégeant au collège départemental consultatif, je regrette aujourd'hui de constater que, semble-t-il, le fléchage de ce fonds reproduit les fractures territoriales. Je souhaiterais disposer d'un état des lieux précis, pour le département de la Seine-Maritime, de ce qui était attribué auparavant par la réserve parlementaire et vers quels territoires et de ce qui est apporté aujourd'hui le Fonds pour le développement de la vie associative. En effet, malgré plusieurs échelons de représentativité au sein des différentes instances consultatives du Fonds pour le développement de la vie associative et la présence de représentants du Parlement, certaines inégalités territoriales semblent persister dans des financements au détriment du monde rural. En tout cas, les chiffres pour 2018 et 2019 le montrent. Il ne s'agit en aucun cas, bien entendu, de priver par ailleurs le tissu urbain et périurbain, qui bénéficie d'un réseau associatif très riche et très dynamique méritant lui aussi d'être soutenu.

d'attribuer aux associations les fonds anciennement versés au titre de la réserve parlementaire, et ce à travers un amendement au projet de loi de finances pour 2018 fixant à 25 millions d'euros les crédits votés à cette finalité. Les mêmes crédits ont été reconduits par les parlementaires lors du vote du projet de loi de finances pour 2019. Aux fins de remplir le nouvel objet de financement de soutien au fonctionnement et aux projets des associations, le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au FDVA a été modifié. Le décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au Fonds pour le développement de la vie associative introduit des principes révisés de répartition des crédits et de gouvernance au plus près du terrain, pour tenir compte des attentes précises exprimées par les parlementaires. En effet, la représentation parlementaire a demandé au Gouvernement que les crédits soient répartis pour moitié de façon totalement égale entre les départements et pour moitié en tenant compte de critères de population et du nombre d'associations dans chaque département. Ce faisant, une plus grande équité territoriale est assurée aux territoires, notamment les territoires ruraux et d'outre-mer. Le décret du 8 juin 2018 a également organisé une gouvernance départementale de l'allocation des subventions allouées par le FDVA, conformément aux attentes des parlementaires. Ainsi, un collège consultatif départemental associe les services de l'État, les collectivités territoriales et les associations, pour la définition des priorités de financement des associations du département comme des propositions de financement. Enfin, ce décret et l'instruction du 15 mai 2018 relative au FDVA et à l'utilisation de ses crédits déconcentrés prévoient que les petites associations sont une priorité L'instruction précise ainsi que les subventions allouées peuvent idéalement s'inscrire dans une fourchette allant de 1 000 à 15 000 euros. Ce faisant, le décret a organisé officiellement les modalités d'attribution de subventions aux associations de métropole et à celles des collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution. Toutes les petites associations de tous les territoires bénéficiant autrefois de la réserve parlementaire ont pu effectuer des demandes de subventions au titre du FDVA pour leur fonctionnement et leurs nouveaux projets, quel que soit leur secteur d'activité, le fonds étant interministériel. En Seine-Maritime, 304 358 euros ont été attribués à 72 associations. À titre de comparaison, en 2016, la réserve parlementaire avait permis de soutenir 162 associations pour un montant de 447 414 euros. Ce département bénéficie donc de 68 % de son ancienne dotation. Dans le cadre du FDVA, et après consultation du collège départemental comprenant des élus locaux, le soutien aux associations en zone rurale a été érigé en priorité de financement de la note d'orientation, notamment en 2019. Deux réunions d'information ont été organisées dans les pays de Bray et de Caux en 2019, et 60 % des associations soutenues dans le département sont de petites associations qui ne sont pas affiliées à un réseau et qui sont exclusivement bénévoles ou s'appuient sur deux salariés au plus. associations implantées en zone de revitalisation rurale ou dans des communes de moins de 1 000 habitants ont bénéficié du FDVA pour un montant de 39 000 euros. Je tiens à votre disposition toutes les précisions relatives au département de la Seine-Maritime.

contre 253 sur le reste du territoire départemental. Cette situation s'est aggravée en 2019 quand on regarde de plus près la répartition

d'un arrêté le 30 décembre 2019 laisse en suspens un certain nombre de questions, notamment au regard de l'interprétation qui a pu en être faite par plusieurs instances qui conseillent les collectivités locales. Selon un article paru sur le site internet de la Banque des territoires le 6 janvier 2020, 2020, « l'État va donc attribuer des ressources à toutes les communes qui justifieront, au titre de l'année scolaire 2019-2020, du fait de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, d'une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire 2018-2019. Il peut s'agir, d'une part, des communes qui ne finançaient pas du tout les écoles maternelles privées, d'autre part, de celles qui les finançaient déjà- soit les deux tiers des communes -et pour lesquelles seule la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire fera l'objet d'une compensation

ceci : « Lors de l'examen de ce projet de décret au Conseil national d'évaluation des normes, le 28 novembre dernier, les représentants des élus avaient soulevé une multitude de problèmes. [ ...] Un certain nombre de questions très concrètes se posent, auxquelles le décret ne répond pas, puisqu'il ne précise pas les modalités d'attribution de l'accompagnement financier selon le type de rapport entretenu par la commune avec l'école maternelle privée. » En conséquence, monsieur le ministre, je souhaite vous poser un certain nombre de questions précises. Je voudrais savoir si ce décret ouvre bien finalement la compensation à toutes les communes, y compris à celles qui participaient déjà sans pour autant verser un forfait à parité, que ce soit ou non une convention. Je voudrais aussi savoir si les communes doivent, si elles souhaitent obtenir une compensation, impérativement verser l'intégralité du forfait dès cette année scolaire et déposer un dossier de demande avant le 30 septembre 2020- j'ai cru comprendre qu'il pourrait même s'agir du 30 septembre 2021 -, ou bien si elles peuvent faire l'objet d'une montée progressive pour le versement de ce forfait, avec un rattrapage des années suivantes. Je voudrais savoir dans quelle mesure un recteur aura la faculté de s'opposer à une demande de compensation exposée par une commune. Enfin, pour les communes qui auraient signé un contrat dit « de Cahors » avec l'État, je souhaite savoir si ces dépenses supplémentaires seront retirées de l'enveloppe normée. La parole est à M. le ministre. Madame la sénatrice est à M. le ministre. Madame la sénatrice Christine Lavarde, à l'occasion des Assises de la maternelle, le Président de la République avait annoncé l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans à compter de la rentrée de 2019. Cette nouvelle donne constitue un moment historique pour tous les enfants. En effet, après l'instauration de la scolarité obligatoire par la loi du 28 mars 1882, seulement deux aménagements ont été pris : en 1936 et en 1959. Cette étape importante s'est traduite dans la loi du 26 juillet 2019 dont l'article 11 instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 6 ans. Cette mesure constitue pour les communes une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. L'article 17 de la loi prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient une augmentation de leurs dépenses obligatoires du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à 3 ans. Par voie réglementaire, le Gouvernement est venu préciser ce cadre d'application. Ainsi, le décret du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 définissent les modalités d'attribution de ces ressources : les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui découlent directement de l'extension de l'instruction obligatoire et qui bénéficieront d'une attribution de ressources de l'État. En ce qui concerne les écoles maternelles privées sous contrat d'association, les communes qui connaissent une augmentation des dépenses de fonctionnement des écoles dans ces conditions et qui n'ont pas donné leur accord au contrat d'association avec l'État pourront bénéficier d'un accompagnement financier de celui-ci. Cet accompagnement concernera aussi, ce doit être très clair, les communes qui participaient déjà aux financements des écoles privées sous contrat sur une base volontaire ou conventionnelle sans pour autant avoir donné leur accord au contrat d'association. Les communes qui avaient donné leur accord au contrat d'association pourront également bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État si leurs effectifs de maternelle ont augmenté, à hauteur des dépenses engagées pour la part d'effectifs supplémentaires. Chaque commune sera donc accompagnée au regard de sa situation créée par la loi nouvelle. En pratique, les communes qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement financier devront adresser leur demande d'attribution de ressources aux services académiques. Cette demande devra être adressée avant le 30 septembre suivant l'année scolaire au titre de laquelle la commune sollicite cette attribution de ressources, après approbation des comptes financiers correspondants, soit, pour l'année scolaire 2019-2020, avant le 30 septembre 2021. Lorsque la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles a été transférée à un EPCI, il appartient à ce dernier d'adresser la demande dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux communes. J'ai demandé aux services académiques d'échanger avec les communes ou les EPCI afin d'identifier, au regard des situations particulières, les dépenses éligibles à une attribution de ressources de la part de l'État et d'évaluer le montant de l'accompagnement financier qui pourra leur être versé. Dans le cadre de ces échanges, les services académiques pourront solliciter, de la part des communes ou des EPCI, diverses pièces justificatives et croiser les données statistiques qui leur auront été communiquées. pourra être demandée par les communes ou les EPCI au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. La procédure de présentation de la demande de réévaluation sera identique à celle qui est prévue pour la demande initiale d'allocation de ressources. S'agissant de l'impact des variations de dépenses ... Merci, monsieur le ministre

Pourtant, ses contours sont souvent encore flous. La loi de 2004 n'appliquait l'interdiction de signes religieux distinctifs qu'aux seuls élèves. En 2013, le Conseil d'État ménageait une exception la non-application de la circulaire dite « Chatel », entérinant l'autorisation effective du port de signes religieux distinctifs par les accompagnants scolaires. En matière de laïcité, les limites du lieu « établissement », du temps « scolaire », et de la fonction « enseignement » ne sont pas toujours claires. La proposition de loi tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation, adoptée au Sénat le 29 octobre 2019, vise à étendre le domaine du lieu. Le domaine du temps est assez bien défini, mais que penser lorsqu'il s'agit du temps de permanence, d'un forum des métiers ou encore de moments plus détendus ? Le domaine de l'enseignement est plus difficile à définir. L'interdiction de port de signes religieux pour les enseignants a été étendue aux élèves enseignants en janvier 2015. Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation a précisé

où une intervenante venue présenter son métier devant une classe de maternelle portait un signe religieux. Bien entendu, les parents n'ont pas apprécié. L'élu s'est alors rapproché de l'inspection académique, qui lui a répondu que cette question relevait de l'appréciation du chef d'établissement. De fait, les chefs d'établissement se retrouvent souvent en porte-à-faux dans ce genre de situation délicate. Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour mieux définir le périmètre de décision des chefs d'établissement confrontés à ces situations particulièrement difficiles ? La parole

unifiée à toute contestation du principe de laïcité, que ce soit dans les enseignements ou dans les moments de vie scolaire, en prenant en compte le statut des différents acteurs. Dans cette perspective, nous avons créé un outil nouveau et très utile, qui est un guide pour les chefs d'établissements : il s'agit du vade-mecum « la laïcité à l'école ». Il est composé de vingt-deux fiches classées en quatre rubriques selon la qualité des personnes concernées par l'application du principe de laïcité : les élèves, les personnels, les parents d'élèves et les intervenants extérieurs. L'approche de chaque situation comporte une analyse juridique et des conseils pédagogiques et éducatifs concrets pour savoir comment réagir et prévenir les atteintes au principe de laïcité. Deux fiches clarifient la question du devoir de neutralité des intervenants extérieurs, qu'ils soient parents d'élèves ou membres d'une association. dans la fiche 22, « port des signes religieux par les parents d'élèves », il est rappelé que les parents d'élèves ont certes un devoir d'exemplarité, mais restent des usagers. Cependant, par un arrêt du 23 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a fait la distinction entre les parents accompagnateurs, non soumis au principe de neutralité, et les parents intervenant dans les classes- qui, eux, doivent arborer une tenue neutre. La fiche 23 traite du cas du port de signes religieux par les intervenants extérieurs non membres de la communauté scolaire. Elle précise que, n'étant pas membres de la communauté éducative, les représentants d'associations ne sont pas contraints au principe de neutralité religieuse. Ce vade-mecum permet une meilleure compréhension du cadre juridique. Il met également en avant l'importance du dialogue entre les différents acteurs en anticipant les difficultés à venir et en mettant en oeuvre avec force et constance une pédagogie de la laïcité. Ce vade-mecum s'inscrit aussi dans un dispositif plus large au service du respect de la laïcité, que ce soit en académie ou au niveau national. Au niveau académique, des équipes « valeurs de la République » sont constituées autour du référent placé auprès du recteur et répondent aux situations et aux interrogations comme aux demandes ponctuelles d'accompagnement. Ainsi, dans le cas que vous avez évoqué, il est possible de solliciter cette cellule pour obtenir la réponse adéquate. Personne ne doit être laissé dans l'expectative sur ces questions. Au niveau national, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a créé une équipe nationale « laïcité et faits religieux » pilotée par la secrétaire générale. Ces équipes sont appuyées par le Conseil des sages de la laïcité que préside Dominique Schnapper et qui a pour objet d'aider et de préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité et de faits religieux, notamment sur des cas inédits. La parole

Or il s'avère que les élèves de certaines zones rurales sont pénalisés par des temps de transport particulièrement longs, qui engendrent beaucoup de fatigue et, logiquement, moins d'heures à consacrer au travail scolaire.

Ces adolescents doivent chaque jour se rendre dans des établissements situés à Beauvais où à Gisors, à une trentaine de kilomètres de chez eux ; ils partent tôt et rentrent tard. La seule solution pour permettre à ces élèves de bénéficier de conditions d'apprentissage optimales serait un meilleur maillage territorial en matière de lycées. Le conseil régional des Hauts-de-France, sensible à cette problématique, a exprimé depuis plusieurs mois sa volonté de construire de nouveaux établissements dans l'Oise. Des réflexions avancées concernent ainsi Grandvilliers et Chaumont-en-Vexin, mais aussi Chambly et Pont-Sainte-Maxence.

un important effort financier de la part de la région, qui a démontré son volontarisme, on ne peut que regretter le flou actuel de l'État. Les élus locaux concernés, mais aussi les parents d'élèves, par ailleurs contribuables, sont légitimement impatients et ne comprennent pas ces atermoiements. Ma question est donc simple

Sur la situation particulière des lycées de l'Oise, des projets et des pistes de réflexion sont en cours- vous l'avez mentionné. Vous avez vous-même été reçu par le secrétaire général adjoint et le directeur de cabinet du recteur au sujet du projet de création d'un lycée à Chaumont-en-Vexin. Le contexte démographique nous impose une réflexion approfondie. Depuis cinq ans, l'académie a perdu 8 568 élèves, dont 1 271 pour le département de l'Oise.

Les projections d'effectifs à cinq ans annoncent également une stabilité du nombre de collégiens. À l'issue du collège, les élèves sont majoritairement scolarisés dans les lycées et lycées professionnels de Beauvais, puis à Gisors dans l'académie de Normandie. Un partenariat entre les deux régions et l'académie de Normandie, concrétisé par la signature d'une convention, a été envisagé. Nous restons ouverts

En ce qui concerne Chambly, on note une stabilité des effectifs sur les cinq dernières années. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la création d'un nouveau lycée sur ce secteur aurait des conséquences importantes sur les lycées déjà existants, qui souffrent d'un déficit d'attractivité.

Je sais bien que l'on ne peut pas prévoir avec une acuité totale les effectifs à venir, mais, à toujours se reposer sur des chiffres qui sont stables, on ne fait jamais rien

placé sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale, est aujourd'hui un acteur de référence dans l'innovation pédagogique, en particulier dans le domaine du numérique éducatif. Il conçoit et édite des ressources ainsi que des services pédagogiques pour accompagner la communauté éducative et propose notamment une offre complète de formations. Ses missions sont notamment de favoriser le développement professionnel des enseignants, mais aussi d'être référent en matière de numérique éducatif. Les acteurs

Avec cette décision, l'avenir du réseau lui-même est remis en cause, alors même que la Cour des comptes a reconnu dans son rapport thématique de juillet 2019 que cet opérateur est un acteur clé du service numérique éducatif.

accompli dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma directeur de la formation continue. Le ministère souhaite affirmer l'identité du réseau Canopé autour de missions pérennes et lui confier un rôle central dans la stratégie ministérielle de renforcement de la formation des personnels en s'appuyant sur une offre de services de haute qualité en matière de formation à distance et de numérique éducatif. Cette ambition renouvelée quant à la participation du réseau Canopé à la mise en oeuvre des priorités ministérielles nous a conduits à ouvrir, dès le mois de janvier 2020, une concertation avec les représentants syndicaux de l'établissement portant sur le recentrage des missions du réseau Canopé et sur l'organisation territoriale de la formation continue. Le premier axe de la concertation permet d'expertiser avec les représentants de l'opérateur les implications d'un repositionnement de Canopé comme opérateur national de la formation continue à distance des personnels. première mission serait de produire des parcours de formation d'excellence pour tous les personnels, plus particulièrement pour les professeurs, les formateurs et les contractuels. Le numérique éducatif constituera une dimension essentielle de l'offre ainsi produite. La deuxième mission du réseau Canopé serait d'assurer la maîtrise d'oeuvre de la production de services et de ressources numériques pour la formation, en veillant à diversifier les formats et à se mettre au standard des meilleures formations en ligne. Sa troisième mission serait le développement et l'animation d'une plateforme de ressources pédagogiques de haute qualité produite par les enseignants eux-mêmes et validée par un processus de démarche qualité.

Il s'agit pour le réseau Canopé d'aider les enseignants à s'approprier un environnement professionnel profondément transformé par le numérique. Les missions liées au service public du numérique éducatif doivent être renforcées, principalement à travers l'objectif de formation de tous les professeurs au numérique et par le numérique.

dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, d'un projet de plateforme de formation initiale en ligne de professeurs doté de 10 millions d'euros- c'est dire l'ambition que nous avons. Le deuxième axe de la concertation vise à optimiser l'articulation territoriale de la formation continue et aboutira

biologique, environnementale, sociale, psychologique. L'éducation nationale assume ce rôle depuis longtemps, car l'école a la responsabilité, en liaison étroite avec les familles, de veiller à la santé et au bien-être des jeunes. En milieu scolaire, la promotion de la santé, inscrite à l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation, est assurée en particulier par l'éducation à la santé. Cette dernière est mise en oeuvre de la maternelle à la classe de terminale au travers d'enseignements transversaux tels que l'éducation à l'alimentation ou encore l'éducation à la sexualité. En référence à la mission émancipatrice de l'école, l'éducation à la santé a pour objectif de contribuer au développement chez les élèves d'attitudes favorables à leur santé et à celle d'autrui et d'approfondir leurs connaissances à l'égard des services de santé et aux évolutions du système de santé. Elle poursuit également l'objectif de renforcer les compétences psychosociales des élèves ; compétences qui favorisent la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Par ailleurs, afin d'inscrire la promotion de la santé dans une approche globale, l'éducation nationale déploie cette année la démarche « école promotrice de santé »- une des mesures concrètes de la stratégie nationale de santé. Cette démarche dynamique et positive inscrit la promotion de la santé au coeur des projets d'école et d'établissement. Elle repose sur l'ensemble des personnels et des partenariats territoriaux et place encore davantage l'élève au centre. En effet, l'école promotrice de la santé renforce l'implication des élèves et l'éducation par les pairs en mettant en place des ambassadeurs santé à partir de la rentrée prochaine. Ces élèves ambassadeurs santé sont des élèves volontaires- deux à quatre élèves par niveau de classe -, qui pourront s'impliquer dans le projet d'école ou d'établissement et transmettre à leurs camarades des messages de prévention par un processus de communication interpersonnelle. En outre, l'éducation nationale veillera à développer chez les élèves un apprentissage de la citoyenneté numérique. Vous l'avez observé, monsieur le sénateur, la gestion des données personnelles sur les plateformes numériques de santé constitue un défi majeur de notre époque. L'école participe à relever ce défi par l'éducation aux médias aux médias et à l'information dès l'école élémentaire. Enfin, l'école ne peut faire tout cela sans l'expertise des partenaires de santé. Ainsi, j'ai demandé au rectorat de se rapprocher des ARS pour déterminer les objectifs de santé publique prioritaires à mettre en oeuvre dans des actions de prévention auprès des jeunes en milieu scolaire. Votre question est donc effectivement d'actualité. Je vous remercie,

Il est difficilement acceptable, pour ne pas dire inacceptable, de voir nos élèves quitter l'école élémentaire sans avoir acquis l'apprentissage de la natation. Certes, il manque des bassins d'apprentissage en France, mais ma question porte sur la formation des maîtres-nageurs sauveteurs En France, on constate une diminution constante du nombre de professionnels formés. Or cette formation exige au minimum une année scolaire à temps plein et coûte 6 000 euros, ce qui explique que, chaque année, les collectivités et les établissements privés ont des difficultés à recruter. Une concertation de dix mois a été menée pour faire ressortir la lourdeur de cette formation des MNS. Pourtant, la solution retenue consiste à allonger la formation de deux à

en cours du soir

C'est pourquoi les enseignants de natation, mais aussi les professeurs des écoles, qui ont aujourd'hui la prérogative d'enseigner, sont nos principaux partenaires métier pour déployer le plan Aisance aquatique national

50 % du temps d'ouverture de l'équipement, alors que ce n'était le cas que pour un petit nombre de mois puisque, pour le reste de l'année, ils devaient être accompagnés par un MNS. Il nous